je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun de vous à observer, au cours j’appelle chacun de vous à observer, au cours de nos échanges, l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.

À ces féminicides recensés, il faut en effet ajouter les 800 tentatives de suicide annuelles de femmes victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques ou de violences répétées.

une femme tous les trois jours qui meurt sous les coups de son compagnon : c’est, en réalité, une femme par jour qui meurt des violences d’un homme. Depuis 2020, le harcèlement moral est une infraction criminelle.

cas qui ont conduit à des condamnations, ce sont le plus souvent les familles qui ont porté plainte. Et que fait on pour le demi millier de femmes qui ont survécu à ces tentatives de suicide ? Les sauve t on, ou attend on une autre tentative de suicide qui, cette fois, sera fatale ?

Le renforcement de la formation des forces de l’ordre, la simplification des démarches des victimes témoignent de notre détermination à protéger chaque femme, partout sur le territoire, et à garantir que justice soit faite.

Ce combat est notamment mené par Yael Mellul, ancienne avocate spécialiste des violences conjugales, qui est venue au ministère ce lundi 25 novembre pour travailler sur le sujet.

Pour autant, malgré cette détermination, les chiffres restent affreusement stables. Je vous ai posé une question précise sur la prévention des suicides des femmes qui ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours. Vous nous avez répondu

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que les réquisitions du procès des viols de Mazan résonnent actuellement dans la salle du tribunal judiciaire d’Avignon, voilà quelques semaines que le monde entier regarde Gisèle Pelicot avec admiration et découvre avec horreur Pourtant, toutes les femmes le savent : si l’ampleur des viols est sans précédent dans cette affaire, le geste, lui, est commun. Ce n’est pas un fait divers ; c’est un fait de société. En 2023, près de 3 millions de femmes ont été victimes de violences sexuelles. Pourtant, seulement 6 % de ces victimes ont porté plainte.

En 2023, le budget de l’État dédié à la lutte contre les violences conjugales s’élevait à 171,7 millions d’euros. Pourtant, selon la Fondation des femmes, ce sont 5,4 milliards d’euros qui devraient être consacrés à la lutte contre ce fléau Rappelons que les violences faites aux femmes nous coûtent, chaque année, quelque 3,9 milliards d’euros. Outre ces investissements financiers indispensables, à quand le retour à un ministère des droits des femmes de plein droit ?

une loi cadre contre les violences sexuelles pour lutter activement contre ces violences systémiques et apporter une réponse visible, cohérente, efficace à ce problème immense

Dans les territoires, les délégations régionales aux droits des femmes sont sous dotées et n’ont pas les moyens de fonctionner. Elles recrutent des jeunes en service civique pour pouvoir assurer des missions de pilotage et de coordination des réseaux. Les associations sont épuisées.

Pendant dix jours, aucune information n’a transpiré sur sa situation. Boualem Sansal a finalement été présenté hier au parquet et placé sous mandat de dépôt pour « atteinte à la sûreté de l’État, à l’intégrité du territoire, à la stabilité ou au fonctionnement normal des institutions, aux symboles de la Nation et de la République ». Il risque, monsieur le ministre, la peine de mort, peine qui sera probablement commuée en prison à perpétuité. Que lui reproche t on ? Probablement de ne jamais avoir trahi sa liberté de penser, sa liberté de dire, notamment ses critiques vis à vis du pouvoir et de l’islamisme, qui gangrène la société. Prix du roman de l’Académie française, est peut être aussi une victime des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, probablement d’ailleurs au même titre que Kamel Daoud, prix Goncourt 2024, interdit de participer au Salon international du livre d’Alger par les mêmes autorités algériennes. L’arrestation de Boualem Sansal est inacceptable, sur la forme, bien sûr, mais également sur le fond, car cet écrivain incarne, pour beaucoup, la promesse d’un avenir loin des lourds héritages du fanatisme et de l’intolérance. Elle est inacceptable, car on s’attaque à un homme qui symbolise, dans ce pays, la défense des droits de l’homme et de la femme. Elle est inacceptable, car c’est la liberté d’expression et la culture que l’on emprisonne. En France, la mobilisation des intellectuels, relayée par les médias de ce côté ci de la Méditerranée, est très importante. Pouvons nous compter, monsieur le ministre, sur une mobilisation aussi forte des autorités politiques et diplomatiques françaises pour venir en aide à notre compatriote ?

de l’écrivain, véritable sentinelle de la liberté. Je veux vous dire, monsieur le sénateur, que rien ne nous permet aujourd’hui d’accréditer les fondements de l’accusation dont il fait l’objet.

Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation des services de l’État pour suivre la situation de Boualem Sansal, qui peut aujourd’hui bénéficier de la protection consulaire à laquelle il a droit en tant que citoyen français. Nous resterons pleinement mobilisés sur ce sujet. Merci de votre engagement, monsieur le sénateur

Comme un écho à cet égoïsme global, la France s’apprête non plus seulement à raboter, mais véritablement à tronçonner son aide publique au développement (APD), de l’ordre d’environ un tiers. C’est la seule mission qui est amputée à ce point De l’euro investi à la tonne de CO2 économisée, en permettant de financer transports publics, énergies renouvelables ou sauvegarde de la forêt en Afrique, cette politique est pourtant notre politique la plus efficace en matière de lutte contre le changement climatique.

Sachant que la politique extérieure de la France est un domaine sinon réservé, du moins partagé, allez vous abandonner le deuxième coup de rabot de 641 millions d’euros prévu par amendement au Sénat, après la baisse déjà massive prévue dans le

je vous remercie de vos questions. Je sais à quel point vous êtes engagé sur ces sujets. Le projet de loi de finances pour 2025 prolonge notre contribution à l’effort collectif engagé cette année. En 2024, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a déjà contribué de façon significative au plan d’économies, avec une réduction de 880 millions d’euros de son budget,

Dans ce cadre contraint, l’effort sur les crédits de l’aide publique au développement devra être réparti sur l’ensemble de nos dispositifs. Nous cherchons à préserver des moyens en faveur de l’aide humanitaire et des outils bilatéraux, qui nous permettent de développer des projets rapides, visible l’action de la France. Nous mettrons tout en œuvre pour défendre nos priorités. Néanmoins, plus généralement, des choix devront nécessairement être opérés, notamment parmi nos engagements multilatéraux. Nous devrons consentir des efforts importants pour absorber cette baisse de crédits dans nos actions multilatérales, notamment dans les domaines du climat, de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de l’égalité entre les femmes et les hommes.

tout est lié. Faisons preuve de responsabilité

En ce triste mois anniversaire des attentats terroristes islamistes sanglants du 13 novembre, alors que la France commémorera bientôt les dix ans des attentats de janvier 2015 et en plein procès Samuel Paty, proposition de loi est particulièrement ignoble. J’imagine l’effroi des victimes du terrorisme islamiste en France et de leurs familles ! Cette initiative a provoqué de vives et légitimes réactions à l’encontre de LFI, qui cherche toujours à faire le buzz, malheureusement rarement pour promouvoir la cohésion et l’apaisement de notre pays et souvent pour le fracturer. Le clientélisme électoral qui sous tend cette proposition de loi ne fait aucun doute. Assigner à résidence une partie de nos concitoyens par le mensonge, le communautarisme, la victimisation et la réécriture de l’histoire est la dangereuse marque de fabrique de LFI. Hélas, il semble que nous ne vivions pas tous dans le même pays ! Alors que nous sommes tous sous la menace permanente du terrorisme islamiste, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, ce texte est une faute. Finalement, monsieur le ministre, cette proposition de loi de la honte nous interroge un parti politique suscitant la haine et le séparatisme ne peut il pas être condamné pour une telle initiative ?

La liberté d’expression ne permet pas tout. Elle ne permet pas de justifier l’injustifiable, notamment les meurtres de nombreuses victimes, commis de façon ignoble.

d’un outil plus opérationnel encore pour lutter contre le terrorisme. Tout retour en arrière serait proprement ignoble et scandaleux. Je ne peux une fois de plus que partager votre émotion. La menace islamiste est toujours très prégnante. Aucun recul

gardant la tête haute, elle a permis d’aider de nombreuses filles et de nombreuses femmes. Oui, il doit y avoir un avant et un après Mazan, un continuum dans la lutte contre le continuum des violences. Nous devons amplifier nos actions. Madame la secrétaire d’État, votre gouvernement a annoncé, ce lundi, de nouvelles mesures, dont l’une porte justement sur la soumission chimique. Les kits de détection seront expérimentés dans certains départements.

quel état des lieux dressez vous avant l’extension du dispositif en métropole et en outre mer ? De janvier à octobre 2024, on dénombre 1 564 victimes de violences intrafamiliales en Finistère, soit sensiblement plus qu’en 2023.

d’abord pour les 330 salariés dont les emplois sont menacés et qui veulent continuer à travailler – des centaines d’emplois indirects pourraient aussi être en danger. Ça l’est ensuite pour l’Aube, où la désindustrialisation a fait tant de mal. Le mythe funeste d’une France sans usines a laissé des plaies béantes, que nous tentons de soigner en conservant nos fleurons sur les territoires, notamment dans le domaine du textile. Enfin, pour la France, le Coq Sportif est une marque iconique. Elle a brillé aux yeux du monde entier lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et nos athlètes ont accompli leurs exploits en arborant le fameux coq tricolore. Cependant, monsieur le ministre, les nuées s’accumulaient déjà à l’horizon depuis bien longtemps. Ainsi, en octobre, l’entreprise annonçait déjà chercher des solutions de financement. Les mauvais résultats de l’an passé se sont malheureusement confirmés au premier trimestre 2024. De façon plus globale, le vent mauvais des fermetures d’usines souffle sur le pays. Il faut poursuivre la dynamique de réindustrialisation dans laquelle le Coq s’est inscrit, y compris en rapatriant son centre de recherche et développement (R&D) en France, non seulement en ouvrant de nouvelles usines, mais aussi en trouvant des solutions de financement et de reprise adaptées. Nous l’avons fait à Romilly, dans la ville du Coq Sportif, grâce au groupe Rebirth, qui vient de reprendre l’usine Cycleurope. Monsieur le ministre, ma question est simple : quel est le plan d’action du Gouvernement pour soutenir le Coq Sportif et préserver notre outil industriel et nos savoir faire ?

durement, ces dernières décennies, par plusieurs vagues de désindustrialisation. Même si, depuis 2016, ce pays crée plus d’emplois industriels qu’il n’en perd, cela n’empêche pas des situations extraordinairement difficiles, comme celle

cotisent à l’assurance chômage dans le pays où ils travaillent, mais qu’ils bénéficient, en cas de perte d’emploi, d’une indemnisation chômage versée par leur pays de résidence. Une compensation entre États est bien évidemment prévue, mais elle est très éloignée des réalités économiques et sociales. Pour l’Unédic, l’indemnisation de ces travailleurs frontaliers représenterait un surcoût de 800 millions d’euros, ce qui dans l’état actuel de nos finances, je le conçois, n’est pas acceptable. Certains de mes collègues ont déjà alerté le Gouvernement sur ce danger : je pense à Annick Jacquemet, ainsi qu’à Cyril Pellevat, qui a récemment déposé une proposition de résolution européenne. Il y a quelques semaines, madame la ministre, vous indiquiez, dans cet hémicycle, que le Gouvernement avait interpellé la présidence du Conseil européen pour avancer sur un nouveau règlement, et qu’il au niveau national en baissant les indemnités et en redéfinissant l’offre raisonnable d’emploi. Je vous propose une troisième voie. Êtes vous prête à entamer sans délai des discussions avec les pays voisins, afin d’aboutir à des accords bilatéraux sur une compensation d’État à État plus juste et plus équilibrée, et, ainsi, à ne pas faire porter l’effort sur les seuls travailleurs frontaliers

Il semblerait qu’Alger cherche de nouveau à nuire à notre pays. On pourrait penser que la cause en est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, mais, en réalité, tous les prétextes sont bons pour attaquer la France. Face à l’expression de cette haine, qui est Boualem Sansal, si ce n’est le bouc émissaire des tensions entre nos deux pays ? Il incarne le courage à travers ce qu’il fait et ce qu’il dit, lui qui, d’une voix longtemps inaudible, a dénoncé les ravages de l’oppression islamiste. Son crime, aux yeux du pouvoir algérien, serait d’être devenu Français et, pire encore, d’aimer la France. L’Algérie s’accommode de son histoire et ne cache pas son mépris envers les juifs, les harkis et, plus largement, les Européens, au premier rang desquels les Français. Que dire des traitements discriminatoires et cruels qu’elle inflige aux Berbères, aux Kabyles, ou encore aux femmes ? Si la France a encore quelque chose à montrer au monde, c’est dans la défense de la liberté et de l’universalisme. Pourtant, sur cette question, nous ne sommes, hélas ! pas unanimes. Une grande partie de la gauche, qui a toujours voulu s’approprier la tradition des Lumières, est totalement muette sur le sort de notre compatriote. Pas ici ! Elle reste plus préoccupée par la suppression du délit d’apologie du terrorisme que par la défense de ce grand écrivain. Plus grave encore, les dérives victimaires de l’Algérie ont trouvé un écho complice dans certains médias du service public. Comment, monsieur le ministre, accepter de tels propos, qui desservent notre pays, qui desservent la démocratie ? Nous parlons de l’emprisonnement arbitraire d’un homme de 75 ans,

qui fait écho à celle du sénateur Demilly, et qui démontre bien l’engagement de l’ensemble de cet hémicycle, ainsi que l’émotion et la stupéfaction de tous les Français à l’annonce de l’inculpation de notre compatriote Boualem Sansal. rappeler ici, une fois de plus, que la France est toujours du côté de l’universalisme, de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion. Aujourd’hui, nous ne voyons rien

de l’État pour suivre cette affaire et faire bénéficier Boualem Sansal des services consulaires auxquels il a droit en tant que citoyen français. Comptez sur la mobilisation de l’État et du Gouvernement sur ce sujet. Et le

Quelle est votre feuille de route ? Sommes nous bien, comme le dit le slogan célèbre, « tous unis contre la vie chère »

Monsieur le ministre, nous assistons depuis plusieurs années à une radicalisation des oppositions face aux projets de retenue d’eau. Nous avons tous en mémoire la violence inouïe des manifestations à Sainte Soline l’an dernier. En Vendée, les dégradations sont de plus en plus régulières. Que ce soit à Nalliers ou à Pouillé en août 2022, ou sur la réserve du Bernard à l’été 2023, le coût des dégradations avoisine à chaque fois le million d’euros. De nombreuses zones sont désormais protégées par des sociétés privées pour éviter les intrusions. Lundi, un nouveau cap a été franchi. À l’Oie, petite commune du bocage, neuf poids lourds et engins de travaux d’une entreprise de travaux publics Un collectif a revendiqué cet acte. Il souhaitait mettre hors d’état de nuire ces machines et menace désormais de s’en prendre aux salariés : « Tout acteur qui s’associera aux futurs chantiers de mégabassines […] en subira les conséquences. » au chef de cette entreprise : il est scandalisé et vit dans la crainte de l’étape d’après. Nous ne sommes pas face à de simples opposants, monsieur le ministre, mais à des groupuscules aux méthodes mafieuses et terroristes, qui n’hésitent plus à s’en prendre directement aux entreprises et à leurs salariés. Dans son communiqué, ce groupuscule mentionne Sainte Soline. De nombreux élus d’extrême gauche n’avaient alors pas condamné la violence inouïe des manifestations. J’espère aujourd’hui que les élus de tous bords s’accorderont unanimement à condamner ces actes odieux et criminels. Monsieur le ministre, nous comptons sur votre fermeté et sur un soutien sans faille de l’État dans la lutte contre ces groupes extrémistes, qui mettent en danger la paix sociale et l’intégrité de nos entreprises et institutions. La parole

ce groupuscule a proféré des menaces et des intimidations vis à vis de l’entreprise et de ses salariés, leur faisant savoir que s’ils devaient se rendre sur un chantier ou une réserve de substitution, il pourrait leur en coûter cher.

bien sûr sous la tutelle de la justice et des procureurs, pour retrouver les coupables. Cela prendra le temps qu’il faudra, mais nous y mettrons les moyens et nous déférerons les responsables devant la justice pour qu’ils soient punis sévèrement. Que les agriculteurs, leurs premières victimes, en soient conscients : nous sommes totalement mobilisés Merci, monsieur le ministre. Nous savons pouvoir compter sur votre engagement. La parole est à Mme Anne Sophie Romagny, pour le groupe Union Centriste.

dans les PME. L’industrie est frappée de plein fouet : il y a deux semaines était annoncée la fermeture de deux usines Michelin dans le Morbihan et en Maine et Loire, ainsi que d’une dizaine de magasins Auchan dans toute la France. Cette semaine, dans le département de la Marne, nous avons appris, en quelques jours seulement, la fermeture du site d’ArcelorMittal à Reims, puis le plan de restructuration du laboratoire Boiron, qui évoque la fermeture de certains sites, dont celui de Reims, et enfin la prononciation de la liquidation judiciaire

Bien sûr, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier : certaines sont en difficulté, mais d’autres, alors qu’elles sont en bonne santé, licencient en raison de choix stratégiques. C’est le cas d’ArcelorMittal.

ne jouent pas le jeu sous le regard de leurs salariés qui perdent leur emploi ? La parole

nationale indiquait que le futur programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle n’était pas figé et que l’idéologie de genre n’était « absolument pas présente dans ce programme ». Monsieur le ministre, un programme était il nécessaire ? Que pensez vous de son contenu ? Assurez vous le Sénat que, dans sa version définitive, le contenu de chaque cycle sera adapté à l’âge des élèves,

Malheureusement, nous vivons aussi une époque où il est interdit d’être spectateur face aux violences sexuelles, en particulier celles que subissent nos adolescents, aux violences intrafamiliales et à la prolifération des images à caractère pornographique dans le quotidien de nos enfants.

rien. Je ne me résous pas à ce que la première image de la sexualité découverte par un gamin le soit dans une cour de récréation, à 9 ou 10 ans, sur le téléphone portable d’un copain. Évidemment, l’école a pour mission de protéger nos enfants et, en même temps, de les aider à construire leur jugement par eux mêmes.

Deuxièmement, le militantisme n’a pas non plus sa place dans notre école. Je veux un encadrement très strict de tous les intervenants

Monsieur le ministre, oui, en ces temps où les enfants sont en permanence exposés, y compris à la pornographie la plus sordide et aux violences conjugales, l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est utile et l’élaboration d’un programme nécessaire. Je suis donc rassuré par vos propos. J’y adhère. J’espère que votre parole portera et que vous serez suivi. Le problème est que, lors de son parcours, ce programme a été malmené par les promoteurs d’une vision qui impose à l’école d’être le remède à tous les maux de notre société,

et surtout, comme vous l’avez dit, ne pas oublier que l’éducation est d’abord et avant tout la mission des parents ! La parole est à M. Rémi Cardon, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. et Républicain. Michelin, Watts, Valeo, la liste est longue, monsieur le Premier ministre. Derrière ces noms d’entreprise, il y a des familles dont le destin est brisé, une angoisse certaine face à l’avenir et un sentiment d’impuissance dangereux. Il s’agit notamment de soudeurs, de chaudronniers, de dessinateurs industriels, d’électriciens, bref, de métiers essentiels dont la noblesse est balayée, alors qu’ils méritent toute notre attention et notre protection. Face à la mondialisation du libre échange à tout va, vous n’avez pas joué votre rôle. Vous avez laissé faire et vous vous êtes laissé faire. Rien ne va : nous sommes en pleine guerre économique avec les États Unis et la Chine, et le solde des ouvertures et fermetures d’usines en France est redevenu négatif

Madame la secrétaire d’État, la convention tripartite relative au fonctionnement de l’université de Corse pour la période 2023 2027 prévoyait une annexe financière consistant en un versement complémentaire à la subvention pour charges de service public de 500 000 euros par an. L’État est donc tenu de verser à l’université de Corse 2,5 millions d’euros sur cinq ans pour couvrir les charges liées à la masse salariale. Pour l’heure, cet engagement n’a pas été respecté.

Cette accréditation est conditionnée à l’octroi de la masse salariale nécessaire, laquelle dépend de la subvention de 500 000 euros que l’État n’a toujours pas versée, ni pour 2023 ni pour 2024. 2024. Pour faire simple, le non respect des dispositions prévues dans l’annexe financière de la convention entrave la mise en œuvre d’un axe pédagogique stratégique, considéré comme prioritaire dans la même convention. Dans une île déjà sous dotée en infrastructures sanitaires – je pense notamment à l’absence de PET scan –, reculer sur les études médicales à l’université de Corte constituerait une régression sans précédent.

Vous m’interrogez sur la question primordiale de l’accès aux soins sur le territoire corse et sur la formation aux études de santé dispensées au sein de l’université de Corse à Corte. Il s’agit d’une question importante, car la Corse doit rester ouverte sur le monde, tout comme le monde est ouvert sur la Corse.

Vous l’avez dit, l’objectif de l’université de Corte est désormais de consolider le premier cycle complet d’études médicales, pour ajouter à la première année déjà existante une deuxième et une troisième année. Sur ce point, un dossier académique est en cours d’examen au sein du ministère. À la suite d’une première expertise, il semble que le dossier de demande d’accréditation doive encore être complété avant son examen par le Cneser.

Soyez assuré, monsieur le sénateur, que le ministère est en lien étroit avec l’université de Corte sur ce sujet. Un temps d’échange est prévu très prochainement afin de préciser certains points du dossier, notamment en ce qui concerne le programme d’enseignement, les conventions avec les établissements de santé ou encore les moyens

portant sur les négociations en cours relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur, en application de

en application de l’article 50 1 de notre Constitution, le Premier ministre a souhaité que soit organisé au Parlement un débat sur l’accord de libre échange entre l’Union européenne et les pays membres

Ce que nous souhaitons, au travers de ce débat, c’est entériner solennellement la position de la France et lui offrir une assise transpartisane forte, pour que la voix de notre pays puisse résonner dans toute l’Europe. Je profite de l’occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant vous pour rassurer nos partenaires d’Amérique latine : nous ne souhaitons pas remettre en cause la relation qui, par sa profondeur historique, unit nos deux continents. Ce que nous souhaitons, en revanche, c’est donner à cette relation l’ambition nécessaire pour qu’elle s’inscrive durablement dans le temps, autrement dit, pour qu’elle se renforce de manière déterminée. Ce constat, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voudrions que nos partenaires européens l’entendent également : la France, les Français ne souhaitent ni la fin des accords commerciaux ni la fin des échanges agricoles. Ces accords ont en effet justement permis à notre pays d’occuper le rang qu’il tient aujourd’hui, celui de sixième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, et de dégager, en 2023, un chiffre d’affaires à l’export de 85 milliards d’euros, ainsi qu’un excédent commercial de 6,5 milliards d’euros. Aussi la France se tient elle pleinement mobilisée pour discuter de nouveaux accords, à la condition toutefois qu’ils s’avèrent favorables aux intérêts français et européens, que les débouchés soient au rendez vous, que nos intérêts essentiels soient pris en compte et que notre modèle agricole et alimentaire soit respecté.

Cette dichotomie, nous le savons, conduit pourtant à compromettre la souveraineté alimentaire des Français et des Européens, au détriment de la qualité de leur alimentation. Aussi, et parce que l’agriculture et l’alimentation sont au cœur de l’identité de notre pays et de notre continent, nous devons signifier aujourd’hui, par notre vote, que nous veillons scrupuleusement à ce que l’agriculture soit traitée à l’international non pas seulement comme un secteur défensif, mais aussi comme un secteur stratégique à promouvoir. Cette ambition, la France la défendra au travers de la promotion des clauses miroirs, qui plus est assorties de contrôles sérieux. En effet, il n’y a pas de raison qu’une norme nécessaire chez nous devienne moins nécessaire quand elle s’applique à un produit importé. Dans le cas contraire, mesdames, messieurs les sénateurs, nous en viendrions à renier les efforts que nous avons consentis, depuis près de soixante dix ans, pour protéger notre modèle agricole européen et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Car c’est bien là tout l’enjeu. Les audits menés depuis 2017 par la Commission européenne le démontrent, les dispositifs d’inspection et de contrôle des pays du Mercosur ne sont pas suffisamment fiables et à même de garantir la traçabilité des produits, et certains des failles qualifiées de systémiques. Dans ces conditions, nous ne pourrions pas garantir à nos concitoyens que la qualité des denrées importées, telle que nous la recherchons en Europe, sera respectée. Nous ne pourrions pas plus assurer à nos agriculteurs que les conditions d’une concurrence loyale seront mises en place. Pour illustrer mon propos, les exemples ne manquent pas. En ratifiant l’accord, nous entérinerions le fait que, dans les 180 000 tonnes de sucre auxquelles le marché européen ouvrirait ses portes, nous pourrions retrouver jusqu’à 145 pesticides, dont nous interdisons pourtant l’emploi en Europe. En ratifiant l’accord, nous accepterions que des aliments qui se retrouveraient dans l’assiette des Européens dépassent jusqu’à six fois les limites maximales de résidus que nous avons adoptées en Europe. En ratifiant l’accord, nous accepterions de retrouver, dans les 180 000 tonnes de volailles supplémentaires qui accéderaient au marché européen, des molécules européen, des molécules déclarées toxiques, mutagènes et cancérogènes, dont nous interdisons légitimement l’usage en Europe. En ratifiant l’accord, nous accepterions donc que les normes de production européennes ne soient pas respectées et que nos agriculteurs se retrouvent

Comme je l’ai dit hier à l’Assemblée nationale, avec cet accord, nous signerions le contrat de délocalisation d’une partie de notre production agricole, car nous importerions, demain, davantage de produits, le respect des normes en moins. Il serait pourtant inacceptable que l’objectif de reconquête de notre souveraineté, que l’Union s’est fixé dans le sillage de la pandémie de covid 19, soit remis en cause pour un secteur aussi vital que l’agriculture.

Aussi, ne laissons pas cet accord, par sa conclusion, rallumer des braises encore mal éteintes, car c’est le lien de confiance qui unit l’Europe et ses citoyens qui s’en trouverait endommagé. et ses citoyens qui s’en trouverait endommagé. La France a donc de sérieuses raisons, concrètes, pragmatiques, de s’opposer à l’accord tel que la Commission l’envisage. L’absence de garanties solides pour nos agriculteurs, notre sécurité sanitaire, notre environnement et notre souveraineté alimentaire préoccupe ailleurs en Europe. Mes déplacements diplomatiques m’ont permis d’en acquérir la conviction. La Pologne – j’ai rencontré son ministre de l’agriculture la semaine dernière – vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle s’opposait à cet accord. sénateurs, si vous en êtes d’accord, le Parlement, le Gouvernement et les Français s’uniront avec détermination, côte à côte, pour convaincre la Commission et les autres États membres

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l’a souhaité le Premier ministre, nous avons aujourd’hui l’occasion d’avoir un débat démocratique sur les négociations relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Ce débat est essentiel, car il était inconcevable, sur une question d’une portée si capitale, de ne pas associer les parlements nationaux. Je m’inscris pleinement dans les propos de ma collègue Annie Genevard et je réaffirme avec force la détermination du Président de la République et du Gouvernement sur ce sujet. Ces négociations, engagées voilà vingt cinq ans, ont été motivées par des intérêts communs, des affinités entre Union européenne et pays du Mercosur, deux ensembles engagés à dialoguer et à commercer pour des raisons géopolitiques légitimes.

Si cette négociation dure depuis plus de vingt ans, ce n’est d’ailleurs pas un argument pour l’achever ; cela prouve justement que quelque chose ne va pas. Nous l’avons rappelé à la Commission européenne, l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur n’est pas qu’un sujet technique. Il a des conséquences majeures pour nos sociétés, nos territoires et nos acteurs économiques. Les agriculteurs, dans la rue, nous le rappellent à leur façon, en construisant des murs avec des parpaings pour représenter la distance qui les sépare de l’administration européenne. La mobilisation remarquable de plus de 600 parlementaires français, qui ont adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, témoigne de l’implication exemplaire de la représentation nationale. Cette force d’engagement nous oblige et nous rappelle que les grandes décisions européennes doivent toujours puiser leur légitimité dans les aspirations et les préoccupations de nos concitoyens. Toutes les opinions doivent être entendues, dans le cadre d’une concertation transparente et démocratique. C’est pourquoi le Gouvernement est pleinement mobilisé pour faire entendre ses positions. À Bruxelles, mardi dernier, j’ai rappelé aux prochains commissaires chargés respectivement du commerce et de l’agriculture notre opposition ferme à la version actuelle de l’accord. Je l’ai redit hier aux représentants des groupes politiques au Parlement de Strasbourg. Mes collègues du Gouvernement et moi même sensibilisons régulièrement nos homologues à travers l’Europe. soyons clairs. La Commission doit respecter le mandat que le Conseil lui a donné. L’accord doit être un accord d’association mixte. Un changement de forme, qui permettrait le contournement du vote à l’unanimité des États membres et de la ratification par les parlements nationaux, serait inacceptable et porterait atteinte au respect des compétences des États membres. Ce serait contraire au mandat de 1999, auquel la Commission ne cesse d’ailleurs de se référer. Le Gouvernement fournit un effort sans précédent pour partager ses préoccupations avec nos partenaires et souligner, à leur attention, le caractère dangereux de cet accord. Ce discours permet de susciter des préoccupations similaires aux nôtres, comme vient de le rappeler la ministre de l’agriculture. La version finale de l’accord n’étant pas encore connue, nombreux sont les États membres qui n’expriment pas encore leur position ; il revient à chacun des États de donner publiquement sa position officielle le moment venu. Il suffit néanmoins d’observer les déclarations publiques de figures majeures de la vie politique dans plusieurs pays européens, tels que la Pologne, ou encore de se référer à l’interview récente de la présidente du Parlement européen pour constater que ce débat est désormais pleinement engagé sur la scène publique européenne et que nombre de nos partenaires partagent

Ce que nous défendons, c’est la qualité de notre agriculture. Ce que nous défendons, c’est la place de nos agriculteurs dans les chaînes de valeur. Ces derniers ne doivent pas être les oubliés de l’histoire commerciale. commerciale. Comme Fernand Braudel dans, nous pouvons affirmer que l’agriculture exprime à elle seule une certaine conception de la France. Elle demeure aujourd’hui l’énergie de nos sociétés, nourrissant les populations, façonnant les paysages et jouant un rôle clé dans la transition écologique. Elle est aussi une activité économique qu’il faut soutenir pleinement. Rappelons le, dans ces moments de bouleversements géopolitiques, défendre l’agriculture n’est pas qu’une question identitaire ou sociale, c’est bien un enjeu stratégique. Ce que nous défendons avec force, c’est notre souveraineté alimentaire, au cœur de la vision de la souveraineté européenne exprimée par le Président de la République à la Sorbonne et à Versailles. Nous voyons émerger une véritable géopolitique de l’alimentation. Des puissances hostiles, comme la Russie, et d’autres peut être demain, instrumentalisent les relations agricoles. Du covid 19 à l’Ukraine, les crises récentes nous rappellent une leçon simple nous ne pouvons pas être dépendants des autres quand notre sécurité est en jeu. Ce que nous défendons également, c’est un monde agricole européen à qui l’on donne les moyens de se battre à armes égales avec ses concurrents internationaux. Souveraineté alimentaire, mais aussi sécurité économique : l’Europe ne peut pas être le dernier dindon de la farce de la mondialisation quand les autres se protègent. Le libre échange, oui, mais avec des critères de réciprocité et de loyauté. Quand on demande à nos agriculteurs et à nos entreprises d’appliquer des normes environnementales ou sanitaires, il est normal de demander à nos partenaires de faire de même et de pouvoir les contrôler. Si le temps agricole est le temps de la terre, il faut aussi protéger le temps long, le cycle des saisons. Or dans sa forme actuelle, cet accord est en décalage avec les défis environnementaux de notre époque. La France s’évertue depuis plusieurs années à défendre une politique commerciale équilibrée et durable. Il y va de la cohérence de nos politiques publiques. Alors que nous imposons à nos producteurs dans tous les secteurs des normes de production de plus en plus exigeantes au nom de l’environnement, nous ne pouvons pas en matière de politique commerciale laisser entrer sur le marché de l’Union européenne des produits moins disants. Ce serait d’ailleurs contradictoire avec le nouveau paradigme que la Commission européenne a elle même défini en 2021 en mettant les enjeux de durabilité au cœur des accords de libre échange. Nous voulons donc que cette approche s’applique pleinement à l’accord entre

suffiraient pas. Il faut que, en cas de méconnaissance de l’accord de Paris par l’une des parties à l’accord UE Mercosur, les bénéfices de ce dernier soient suspendus pour la partie fautive. Nous n’acceptons pas davantage un accord dont les dispositions en matière de développement durable seraient dépourvues de force exécutoire, c’est à dire d’un dispositif de sanction. Nous ne sommes pas seuls à partager ces convictions. De nombreux États sont très inquiets des conséquences environnementales et agricoles de cet accord et sont susceptibles d’exprimer avec nous des demandes additionnelles pour protéger nos filières. Pour notre part, nous estimons qu’il faut rééquilibrer l’accord de manière importante en y ajoutant des conditions additionnelles robustes concernant l’environnement et l’accord de Paris, d’une part, et un mécanisme de sauvegarde particulièrement protecteur dans le domaine agricole, d’autre part.

Le projet d’accord commercial avec le Mercosur nous place en situation défensive et ce n’est pas acceptable. Cela ne signifie nullement que la France et le Gouvernement souhaitent que l’Europe se replie sur elle même et se ferme au commerce. L’Europe et la France sont des grandes puissances exportatrices ; nos agriculteurs, qui exportent l’excellence française au delà de nos frontières, le savent mieux que quiconque ! Dans le domaine industriel, nous avons besoin d’accords de commerce pour continuer de diversifier nos approvisionnements, d’ouvrir de nouveaux débouchés et d’accompagner nos entreprises dans la sécurisation de leurs relations d’affaires.

C’est pourquoi nous devons signer des accords commerciaux répondant à nos intérêts stratégiques réciproques. Plusieurs exemples récents nous montrent que c’est possible : je pense à l’accord UE Chili, améliorant l’accès au lithium, ou encore l’accord UE Nouvelle Zélande sur l’écologie. De tels accords, complets, équilibrés et politiques peuvent alors être des outils géopolitiques puissants. Oui, l’Union européenne doit nouer des partenariats internationaux à travers le monde. Oui, les pays du Mercosur sont des pays avec lesquels nous partageons une communauté de valeurs, des intérêts économiques et géostratégiques importants. Du reste, le Président de la République l’a rappelé avec conviction lors de son récent déplacement en Argentine et au Brésil : le lien qui unit l’Europe et l’Amérique latine est fondamental,

protéger nos intérêts, comme les autres n’hésitent pas à le faire sur le reste de la planète, et le modèle de société que nous défendons au nom de nos préférences collectives. Il s’agit là de trois points essentiels, non négociables Depuis cette tribune, je tiens à vous assurer de ma détermination absolue et de celle de l’ensemble du Gouvernement à marteler notre position et à partager nos arguments de bon sens avec nos partenaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, votre voix compte ; elle est même cruciale. Vous allez voter sur la déclaration du Gouvernement, qui propose de s’opposer à l’accord UE Mercosur tel que la Commission européenne l’envisage aujourd’hui. Votre mobilisation constante est entendue à travers toute l’Europe, notamment par vos collègues parlementaires européens. Vous êtes des acteurs clés de ce combat. La diplomatie parlementaire en direction de vos homologues de tous les pays européens et vos relais à Strasbourg et à Bruxelles sont des leviers puissants pour porter nos préoccupations et nos exigences au plus haut niveau. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui afin de nous prononcer, à la demande du Gouvernement, sur l’accord l’accord négocié par la Commission européenne avec les pays du Mercosur. Cette situation est inédite à plusieurs titres et doit nous pousser à une réflexion collective sur le processus qui nous y a amenés.

inédite, parce que, en lieu et place du large assentiment qu’il devrait recevoir, il fait sur nos travées l’unanimité contre lui. Elle est enfin inédite par le danger que fait peser cet accord sur notre souveraineté alimentaire et l’incompréhension qu’il susciterait dans le monde agricole. Depuis son arrivée à la tête de la Commission européenne en 2019, Mme von der Leyen proclame que la politique commerciale doit entrer dans une nouvelle ère et qu’elle souhaite incarner une Commission « géopolitique Nous ne saurions mieux demander. Nos concitoyens ont depuis longtemps constaté par eux mêmes certains effets néfastes de la politique commerciale pratiquée par la Commission Pour autant, le monde n’est plus celui d’il y a vingt cinq ans. La compétition internationale s’est intensifiée. Les acteurs se sont multipliés, de nouvelles puissances ont émergé. D’autres enjeux, les questions environnementales en tête, sont venus s’ajouter à l’équation. Nous n’avons pas aujourd’hui le même recul sur le libre échange qu’en 1999. De fait, la politique commerciale commune, l’un des piliers de la construction européenne, doit, elle aussi, évoluer radicalement. La puissance commerciale que représente l’Union européenne doit nous permettre de corriger les défauts de ce type d’accord. Il est l’heure pour l’Europe de mettre fin aux dépendances qui affectent sa souveraineté, de sortir de la naïveté dans laquelle elle s’est réfugiée et enfin de défendre résolument les intérêts des Européens, des consommateurs, de nos entrepreneurs, de nos industries et de notre agriculture. de la Commission européenne tente de nous présenter cet accord comme une victoire du libre échange. C’est plutôt un coup de massue donnée au monde agricole, en totale contradiction avec ce que l’Europe impose à ses propres agriculteurs depuis de nombreuses années. À l’heure où le verdissement de la politique agricole commune et le engagent notre agriculture dans une transition à marche forcée, comment comprendre les initiatives qui déstabiliseront nécessairement l’outil de production, affaiblissant davantage encore notre souveraineté alimentaire ? Les agriculteurs subissent déjà les effets de la surtransposition des normes européennes et la chute de compétitivité qui l’accompagne. Cette tradition, typiquement française, nous condamnera demain à ne plus être acteurs de notre consommation. Le projet d’accord n’est évidemment pas sans vertu des secteurs et des industries européens, comme la chimie, l’automobile, le secteur pharmaceutique, bénéficieraient de nouvelles opportunités offertes par l’accord de la compétition internationale, face aux tensions géopolitiques qui perturbent toujours plus les chaînes de valeurs, il apparaît nécessaire de chercher à sécuriser nos approvisionnements stratégiques, notamment en matériaux critiques. Songeons ainsi qu’il y a vingt ans l’Europe pesait encore 30 % de la production mondiale, alors que, d’ici à 2050, sa part sera tombée sous les 10 %. Gardons enfin en tête

de renoncer à une politique de concurrence fondée sur un principe aussi simple que celui de la réciprocité ? Je le redis avec force : l’agriculture n’est pas une activité comme les autres, elle est un pilier de notre existence ! Après des décennies de prospérité, nous avons parfois tendance à oublier la place centrale de l’enjeu alimentaire. Tous les travaux de prospective le soulignent : il redeviendra chaque jour plus fondamental au cours de ce siècle. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs de notre pays nous envoient un signal d’alarme sur leurs difficultés à exercer et à vivre de leur travail. Nous entendons leur appel et devons leur apporter des réponses concrètes et immédiates. Pour cela, madame la ministre, nous comptons sur votre détermination et sur celle du Gouvernement afin d’avancer rapidement dans les prochaines semaines.

Dans l’ombre des discours sur la compétitivité, ce sont le monde agricole dans son ensemble et les consommateurs qui paieront le prix fort de cet accord ! En effet, nos industries et nos agriculteurs sont confrontés à toujours plus de normes, au nom de la nécessaire lutte contre le changement climatique, afin non seulement de protéger la santé de nos concitoyens, mais aussi d’assurer le bien être animal. Comment pourrions nous alors importer des produits qui ne respectent pas ces normes ? Comment tolérer que nous imposions à nos éleveurs de volailles de réduire la taille de leurs élevages pour ensuite autoriser les volailles de fermes usines brésiliennes ? Comment accepter que nous demandions à nos éleveurs de viandes bovines de maintenir un élevage en pâturage pour ensuite avaliser l’import de viandes engraissées aux antibiotiques de croissance ? Comment pourrions nous interdire toute une série de pesticides à nos céréaliers, tout en approuvant du maïs brésilien traité par des produits interdits depuis plus de vingt ans en France La Commission européenne assure qu’elle veillera au respect des normes sanitaires européennes pour l’importation des produits venant du Mercosur. Comment répondre à cette exigence sans mettre en place de véritables clauses miroirs ? De même, comment ne pas être inquiet lorsque l’on connaît l’insuffisance des moyens

garder à l’esprit les volumes que le Mercosur est capable de fournir dans ses secteurs de prédilection. Ils sont immenses ! Les quotas préférentiels que nous lui octroierons seront donc non seulement remplis, mais ils pourraient en outre stimuler encore davantage les filières d’exportation qui existent déjà vers l’Europe.

qui n’est pas au rendez vous des attentes des agriculteurs, sait que cet accord ouvre la porte à une concurrence déloyale. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre vote aujourd’hui réaffirmera notre engagement envers les agriculteurs pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions et pour empêcher la signature d’un accord mortifère pour notre souveraineté alimentaire. Notre vote enverra également un message à destination de la Commission européenne, un message d’unité transpartisan des deux assemblées. C’est un point suffisamment rare dans notre pays pour être relevé, en particulier dans le contexte politique que nous connaissons. Dès lors, apparaît inconcevable que cet accord entre en vigueur contre la volonté de la France, seconde économie et première puissance agricole européenne. Les traités européens sont très clairs, le mandat de négociation donné à la Commission européenne est encore doit être ratifié à l’unanimité des États membres. Je tiens sur ce point à rappeler qu’en début d’année le Président de la République s’était réjoui d’avoir réussi à suspendre les négociations en cours comme la France le demandait. Pourtant,

consistant à scinder ceux ci afin d’en mettre en œuvre les dispositions en se contentant de la majorité qualifiée, est inconcevable. Sur un sujet d’une telle importance, balayer d’un revers de main l’avis de la France, celui de sa représentation nationale, aurait donc nécessairement de profondes conséquences politiques. L’exigence démocratique doit désormais conduire les autorités européennes, comme les gouvernements d’ailleurs, à associer beaucoup plus étroitement les Parlements nationaux au processus de négociation des accords. Madame la ministre, monsieur le ministre, le Gouvernement doit continuer de s’opposer, avec toujours plus de fermeté, à cette manœuvre de la Commission européenne. Il doit en parallèle s’assurer d’amener davantage de partenaires européens à suivre notre position. À cet égard, nous nous réjouissons

parlementaires rejoignent la position française. Mes chers collègues, aujourd’hui, nous réaffirmons collectivement que l’agriculture tient une place centrale dans notre société et qu’elle représente bien plus que l’image d’Épinal à laquelle bien souvent. L’agriculture irrigue chacun de nos territoires, contribue au développement économique et à l’aménagement du territoire. Elle est à l’origine de traditions et de savoir faire millénaires. est enfin le premier acteur de la transition écologique et la première victime du changement climatique. Nous restons convaincus que ces accords peuvent être un relais de croissance puissant, un stimulant économique nécessaire et un outil diplomatique et stratégique fondamental pour la souveraineté de notre continent face aux tendances lourdes qui nous traversent. En revanche, nous refusons avec fermeté un accord qui donne une prime à la concurrence déloyale sur nos marchés, qui va à l’encontre de tout ce que nous faisons pour protéger et améliorer le travail de nos agriculteurs et qui, finalement, emportera avec lui ce qu’il reste de notre souveraineté alimentaire.

Je m’inquiète d’ailleurs de la signification du vote que vous nous demandez, n’ayant reçu aucune proposition écrite d’une éventuelle communication ou résolution. S’agit il d’un soutien au Gouvernement, d’une adresse à la Commission européenne ou d’une rupture stratégique ? nous ne souhaitons pas nous retrouver dans le rôle de l’idiot utile et nous vous invitons à vous souvenir à l’avenir du rôle du Parlement pour discuter des politiques et des positions que la France défendra au Conseil.

Que s’est il passé depuis l’accord avorté de 2019 ? Rien ! Le compte n’y était pas ; il ne l’est toujours pas. Rien, sinon que la France se trouve aujourd’hui isolée, comme en atteste sa perte d’influence en Europe.

Rien, sinon que le Gouvernement a soutenu le report du règlement sur la déforestation, ouvrant ainsi une brèche dans l’accord et les négociations, et que le Président de la République a sonné le premier la charge contre la réglementation verte en Europe.

que la guerre commerciale entre la Chine et le reste du monde s’intensifie, que le multilatéralisme est en panne, à l’image de la paralysie de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et que nous connaissons une guerre d’agression à nos portes. ans que l’Union européenne dispose d’un mandat de négociation totalement obsolète, que les problèmes de fond posés par l’accord de 2019 sont connus et restent d’actualité. Tout d’abord, cet accord est dangereux pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Le fossé entre le cadre réglementaire européen et la pratique dans les pays du Mercosur sur les normes environnementales, sanitaires et de bien être animal représente un double risque, économique pour nos agriculteurs, soumis à une concurrence déloyale, et sanitaire pour les consommateurs européens. Alors que l’Union européenne a acté des positions ambitieuses pour faire évoluer notre agriculture, avec le Pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, autoriser aujourd’hui des produits ne respectant pas nos normes serait un terrible désaveu pour nos agriculteurs, qui n’ont comme ambition que de nous nourrir sainement. Ainsi, la quantité de pesticides utilisés au Brésil est deux fois plus importante qu’en France et 145 d’entre eux sont interdits en Europe, car dangereux et cancérigènes. Les limites maximales de résidus sont dans la plupart des cas plus élevées que ce qu’autorisent les normes européennes. De même, les activateurs de croissance et les antibiotiques sont largement répandus dans l’élevage. Madame la ministre, monsieur le ministre, il n’est pas acceptable que l’Union européenne ouvre 180 000 tonnes de nouveaux quotas d’importation de viande de volaille à droits de douane nuls, élevés dans des fermes usines cinquante fois plus grandes que les exploitations autorisées en Europe, alors que la moitié des poulets que nous consommons sont déjà importés. Il n’est pas acceptable que l’Union européenne, qui encourage le pâturage sur nos territoires, accepte l’entrée de 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaires, engraissée aux antibiotiques dans des exploitations de plus de 10 000 têtes, qui s’ajoutent au cumul des milliers de tonnes déjà autorisées dans les autres accords. Il n’est pas acceptable d’autoriser l’importation d’un million de tonnes supplémentaires de maïs chaque année, à zéro droit de douane, traité à l’atrazine, herbicide interdit depuis plus de vingt ans en France, alors que nos agriculteurs réduisent l’utilisation de pesticides. Il en va de même pour l’ouverture de quotas additionnels sans droits de douane pour le sucre, qui déstabiliseraient nos filières ultramarines, ou encore l’éthanol. Tout cela n’est pas acceptable Alors que l’Europe se fixe des ambitions élevées et s’impose des conditions strictes de production, l’arrivée de ces produits sur nos marchés se fera au détriment des producteurs et éleveurs européens sur fond de distorsion de concurrence, de pression sur les prix et d’absence de contrôle. Au delà des volumes, ce sont aussi les conditions de production des pays du Mercosur qui alimentent les inquiétudes. Ainsi, le Brésil a récemment suspendu ses exportations de viande de génisses à la suite de l’un des trop rares audits de la Commission européenne sur place. démontré que les autorités locales n’étaient pas en mesure de vérifier que ces produits ne contenaient pas de trace d’une hormone de croissance, l’estradiol 17 ß, interdite dans l’Union européenne depuis 1996, attestant de l’impossibilité d’avoir confiance dans le système de traçabilité brésilien. Plus largement, cet accord ferait peser un risque majeur sur la sécurité des approvisionnements agricoles et de leur traçabilité alimentaire, portant atteinte à notre souveraineté alimentaire et à la bonne information des consommateurs. Au Brésil, l’aboutissement de cet accord profiterait essentiellement aux immenses exploitations agricoles qui produisent sans aucune considération environnementale et sociale, au détriment des petits producteurs qui n’auront pas les moyens de résister à la pression sur les prix et aux peuples autochtones chassés de leurs terres. Alors que certains acteurs sud américains commencent à douter de l’intérêt de cet accord, celui ci pourrait bien être perdant perdant, en n’apportant pas les bénéfices promis aux pays du Mercosur et en les forçant à poursuivre un modèle de production intenable du point de vue environnemental

Cette déforestation, principalement liée à l’élevage et à la production de soja, contribue massivement aux émissions de gaz à effet de serre et à l’effondrement de la biodiversité. Alors que l’Union européenne a adopté un règlement pour lutter contre les produits issus de la déforestation, que la droite européenne cherche malheureusement à affaiblir, ratifier cet accord serait un non sens législatif et historique, totalement incompatible avec le respect de l’accord de Paris. Cet accord est néfaste pour le climat, néfaste pour notre souveraineté alimentaire, néfaste pour la qualité de ce que nous consommons. Il est dangereux pour nos agriculteurs : tel est le message qu’ils vous adressent par leur mobilisation, madame la ministre, monsieur le ministre,

Alors que nos agriculteurs font des efforts pour satisfaire les nouvelles exigences de la société, ce qui entraîne des coûts importants et suppose des transitions parfois difficiles, ce dispositif financera inévitablement la disparition de pans entiers de nos sociétés en achetant le silence des derniers agriculteurs français et européens Très concrètement, madame la ministre, monsieur le ministre, l’agriculture ne doit pas être la variable d’ajustement des intérêts offensifs des États membres. Elle n’est pas un objet de marchandage. Il ne peut pas y avoir de entre malbouffe et belles voitures. Céder, c’est renoncer à nos ambitions. Nous demandons depuis de nombreuses années une réorientation radicale de ces accords, qui doivent être des outils au service de nos intérêts stratégiques. La force de l’Union européenne réside dans sa capacité de régulation. Elle seule peut défendre aujourd’hui un modèle de développement durable en utilisant la puissance de son marché intérieur. Nos accords doivent redevenir de réels partenariats économiques et politiques, fondés sur la défense des droits humains, le respect des objectifs de développement durable de l’ONU, de l’accord de Paris, de la protection de normes sociales et environnementales élevées. Ils devront intégrer des clauses de réciprocité des normes, des clauses miroirs, des mécanismes contraignants assortis de sanctions et des clauses de revoyure assurant un réel contrôle démocratique. Ils devront également comporter des clauses de devoir de vigilance et de responsabilité sociétale des entreprises des pays concernés. Le culte du libre échange, qui a transformé l’Europe en continent de consommateurs dépendant de ses concurrents et qui a conduit à une casse sociale d’ampleur dans nos régions, favorisant au passage la montée des souverainistes et de l’extrême droite, ne doit pas aujourd’hui détruire la cohésion européenne. En cédant à des intérêts économiques immédiats, l’Europe se mettrait en danger, en exposant ses divisions internes sur des intérêts offensifs divergents, risquant de compromettre l’unité nécessaire pour défendre une vision commune. L’Europe s’affaiblit sur la scène internationale et pourrait, si nous n’y prenons garde, être empêchée de défendre ses principes de durabilité et de solidarité. Nos concitoyens, quant à eux, manifestent une défiance persistante à l’égard de cet accord. La crise de confiance est nourrie par la Commission européenne, qui poursuit tambour battant les négociations de nouveaux accords tous azimuts, dans une logique purement libérale. Et bien qu’ayant reçu un mandat pour négocier un accord mixte, l’Union européenne envisage de scinder l’accord en deux et de faire adopter ses dispositions commerciales à l’encontre du mandat donné par les États, ce qui poserait un problème de légitimité démocratique. Les résolutions adoptées à l’Assemblée nationale en 2023 et au Sénat en 2024 ont déjà souligné que les conditions démocratiques, économiques, environnementales et sociales n’étaient pas réunies pour signer cet accord. Vous avez donc, madame la ministre, monsieur le ministre, un large soutien de l’opinion publique et des parlementaires. Mais qu’en ferez vous ? Un message à la Commission pour rappeler que vous ne voulez pas de cet accord en l’état ? Un appui pour trouver une minorité de blocage, aujourd’hui difficile à constituer ? Madame la ministre, monsieur le ministre, nous vous soutiendrons, mais ce mais ce que nous vous demandons, au delà, c’est d’obtenir un moratoire sur l’ensemble des accords commerciaux en cours ; c’est de repenser notre modèle d’échanges commerciaux, de replacer la légitimité démocratique en son centre et d’agir pour des accords ambitieux et respectueux socialement et environnementalement.

nous sommes aujourd’hui réunis pour débattre de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Pour la troisième fois, nous allons collectivement exprimer notre opposition à la ratification de cet accord en l’état, proposée par la Commission La Pologne a hier officialisé son opposition à cet accord, s’alignant ainsi sur les positions françaises. Permettez moi tout d’abord de saluer l’engagement personnel du Premier ministre Michel Barnier et de son gouvernement, afin de convaincre d’autres pays européens pour constituer une indispensable minorité de blocage. Le contexte est aujourd’hui inflammable ; c’est peu de le dire. D’une part, la présidente reconduite de la Commission européenne souhaite accélérer la finalisation d’un accord d’hier, pour ne pas dire d’avant hier, au risque d’un passage en force institutionnel. D’autre part, alors même que le deuxième acte des contestations agricoles s’intensifie sur nos territoires, il nous faut aujourd’hui avoir à l’esprit que 76 % des Français s’opposent à cet accord. Notre débat d’aujourd’hui est plus que nécessaire. Rappelons que, pour les pays d’Amérique latine, l’Europe a fait figure de modèle d’organisation. En effet, le rapprochement initial entre les pays d’origine du Mercosur s’inspire de l’expérience de la construction européenne. Comme l’a dernièrement indiqué la ministre Sophie Primas, le Brésil est le premier partenaire commercial de la France en Amérique latine. Nous n’avons donc pas attendu le Mercosur. Dans ce débat, il est nécessaire de souligner que nous ne remettons nullement en cause le principe d’une relation plus approfondie entre les pays de l’Union européenne et ceux du Mercosur. Mais le groupe de l’Union Centriste tient à rappeler trois lignes de force. Première ligne de force, protection n’est pas synonyme de protectionnisme. Le retour d’un isolationnisme américain et de l’agressivité commerciale chinoise oblige l’Europe à s’organiser et à réagir sans naïveté. Dans ce désordre international, elle a besoin d’alliés. Le rapprochement avec les pays d’Amérique latine, d’Amérique du Sud, peut alors ouvrir des possibilités, notamment économiques, mais notre préoccupation porte sur les déséquilibres commerciaux que peut créer l’accord dans sa forme actuelle. En 2017, l’Union européenne connaissait avec le Mercosur une balance commerciale déficitaire de 20 milliards d’euros sur les produits alimentaires et légèrement excédentaire sur les produits industriels. Aujourd’hui, nous craignons que ce déséquilibre préexistant ne s’accentue. Une étude d’impact menée par une université britannique a confirmé l’aggravation du déséquilibre actuel, une baisse anticipée de la production agricole

des accords commerciaux, alors que la Commission européenne elle même imagine un fonds de compensation pour dédommager nos agriculteurs. C’est inacceptable et inenvisageable Alors que l’impératif de souveraineté alimentaire s’est inscrit à notre agenda, les agriculteurs ne demandent pas la charité ; ils défendent un projet d’entreprise et souhaitent pouvoir vivre dignement de leur activité. C’est un engagement de beaucoup d’entre nous dans cet hémicycle. Voilà qui rejoint notre deuxième ligne de force : le pragmatisme ne doit pas céder à la caricature. Le projet d’accord ne peut pas être le bouc émissaire d’une agriculture européenne en proie à des difficultés, faute de choix stratégiques. Si le compte n’y est pas pour certaines filières, d’autres peuvent malgré tout y trouver un intérêt. Je pense notamment à l’automobile, au vin ou encore à l’approvisionnement en métaux rares. Comment ne pas souhaiter une meilleure reconnaissance de nos produits, de nos labels, de nos appellations d’origine contrôlée ? Mais comment ne pas partager l’incompréhension des agriculteurs, à qui l’on demande d’être toujours plus vertueux tout en ouvrant nos frontières à des produits qui ne respectent pas nos normes européennes ? Si le contingent négocié ne constitue pas le raz de marée annoncé, il peut néanmoins déstabiliser nos filières, poussant les prix à la baisse. Le rapport rendu en 2020 par une commission indépendante présidée par Stefan Ambec parle à juste titre d’une « occasion manquée » pour l’Union européenne d’obtenir des garanties environnementales et sanitaires. D’autant que, depuis la signature du volet commercial de l’accord en 2019, les ambitions environnementales des politiques européennes ont été rehaussées par la précédente commission. Elles sont d’ailleurs un des catalyseurs de la crise actuelle. Comment peut on imaginer que la présidente von der Leyen, qui a promu la stratégie, avec son lot de contraintes réglementaires et ses conséquences sur l’agriculture européenne, ait si peu d’exigences dans cet accord sur la qualité environnementale, sanitaire et normative des importations ? de notre troisième ligne de force : fervents Européens, nous pensons qu’il faut donner une place accrue au contrôle démocratique de ces accords commerciaux. Il nous semble important de souligner que le Parlement européen a rappelé à plusieurs reprises, en 2018 notamment, le caractère mixte de cet accord, donc la nécessité d’une ratification à l’unanimité par les parlements nationaux. Le politologue bulgare Ivan Krastev parle de « démocratie frustrée quand la mondialisation, auparavant présentée comme un jeu à somme positive, creuse les inégalités, faute de vigilance démocratique. La première des exigences est la convergence réglementaire. Il n’est pas acceptable d’exonérer nos partenaires commerciaux de contraintes que nous imposons à nos acteurs économiques. Il nous semble donc que des clauses miroirs couplées à des moyens de contrôle sont nécessaires. Une simple annexe ne saurait en effet compenser le manquement constaté du volet commercial. La deuxième des exigences est la transparence des négociations. Nos concitoyens et les parlements nationaux sont en droit de mieux connaître les enjeux de cette nouvelle génération d’accords, qui va au delà de simples aspects commerciaux. Et la troisième exigence est la responsabilité. Les parlements nationaux doivent être davantage associés dans les négociations et dans leurs évaluations. Nous partons, je le crois, L’exécutif européen doit s’attacher à la protection de nos standards, alors même que, à titre d’exemple, l’audit mené au mois d’octobre dernier par la direction générale de la santé de la Commission européenne illustre la défaillance du système de contrôle brésilien de la grippe aviaire.

ni à notre époque, ni à nos ambitions actuelles, ni même à la situation géopolitique à laquelle nous sommes confrontés. De plus, il fait peser un risque beaucoup trop important sur notre souveraineté alimentaire. Il va à l’encontre des grands principes que nous nous imposons à nous mêmes. Or, la réciprocité est aujourd’hui indispensable pour rapprocher nos deux continents et rassurer nos concitoyens européens. Madame la ministre, monsieur le ministre, pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de la déclaration du Gouvernement et s’oppose fermement en l’état à l’état à la ratification du Mercosur ainsi proposé par la Commission. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, et compte tenu de l’unanimité assez rare qui règne sur le sujet, nous n’éviterons pas les redites. Mais ce qui compte, c’est l’unité de la Nation face à ce péril, qui nous menace tous. Nous ne pouvons pas, madame la ministre, monsieur le ministre, demander à nos agriculteurs de respecter des normes et à nos industriels d’œuvrer à la décarbonation de leurs activités dans le même temps des droits de douane sur les biens qui ne respecteraient pas ces règles. C’est pourtant cette position schizophrénique que nous demande d’accepter la Commission européenne sur l’accord J’ai entendu les positions de chacun, mais je rappelle ici que le Président de la République a pourtant été clair à maintes reprises : « […] cet accord tel qu’il a été conçu et pensé, ne peut pas être compatible avec notre agenda climatique et de biodiversité Cette phrase, prononcée en 2021, témoigne que la France n’a pas attendu ces derniers mois pour s’opposer à cet accord. Alors que certains médias et oppositions cherchent une nouvelle fois à rompre l’unité nationale que nous devons avoir en la matière, je tiens à rappeler que le président de la République a toujours et invariablement défendu la position française celle d’un refus clair et sans tergiversation de l’accord tel qu’il est aujourd’hui présenté par la Commission européenne. La France se bat chaque jour dans les négociations pour protéger les secteurs qui risquent de pâtir de l’accord, notamment certaines de nos filières agricoles et alimentaires. Nous ne transigerons pas sur le respect de nos normes environnementales et sanitaires, comme sur la mise en œuvre effective de l’accord de Paris sur le climat. Sur ce dernier point, nous faisons face à un blocage supplémentaire : l’Organisation mondiale du commerce. Elle n’utilise pas l’accord de Paris dans les accords de libre échange. La solution paraît alors toute trouvée. Il suffirait que cet accord sur le climat soit transcrit par l’OMC. De la sorte, il ferait partie intégrante des accords commerciaux dans le monde. Or, ni la Chine, ni les pays du Mercosur, ni – et encore moins – les États Unis, avec le retour de Donald Trump au pouvoir, ne veulent de cette retranscription, source d’une modification profonde du commerce mondial et de son fonctionnement actuel. Pourtant, pouvons clairement pas accepter que 99 000 tonnes de bœufs, 180 000 tonnes de volailles et 25 000 tonnes de porcs par an entrent en Europe à un taux préférentiel de 7,5 %, contre 40 % aujourd’hui, sans respecter les normes européennes – cela a déjà été souligné à maintes reprises – qui s’appliquent à nos agriculteurs. Reconnue pour son excellence, notre production se distingue par sa fiabilité, grâce à la qualité, notamment sanitaire et environnementale, de nos exploitations et à la stabilité de leur rendement. l’accord avec le Mercosur, nous créerons automatiquement une concurrence déloyale pour nos éleveurs, mettant en danger l’agriculture française, qui fait notre fierté et garantit notre souveraineté alimentaire. En défense, la Commission européenne argue que ces produits importés ne seraient pas de nature à déstabiliser les filières européennes, car ils ne représenteraient que 1,6 % de la production européenne, atténuant le risque économique pour les éleveurs. Elle oublie de dire que les accords de libre échange, y compris le Mercosur, ne portent que sur des pièces nobles de la carcasse, les filets, les faux filets ou encore l’entrecôte, que les marchés européens peinent déjà à absorber. Depuis une vingtaine d’années, les habitudes ont en effet évolué vers une plus grande consommation de viande hachée au détriment des pièces nobles. C’est vrai en Europe, mais également aux États Unis et en Amérique du Sud. Ainsi, les pays du Mercosur ont, eux aussi, une consommation principalement axée sur la viande hachée et préfèrent exporter en Europe leurs pièces nobles à haute valeur ajoutée, leur permettant de marger plus sur leurs exportations. La conséquence pour les éleveurs européens est colossale. Contrairement à ce qui nous est annoncé – un taux de 1,6 % –, les pièces exportées dans tous les accords de libre échange cumulés, en y ajoutant le Mercosur, représenteraient 25 % de la consommation des pièces nobles en Europe. Cette concurrence directe et déloyale enlèverait définitivement toute compétitivité aux éleveurs français et européens. À terme, nous risquons la disparition de nos productions, au profit d’une consommation de produits importés aux normes sanitaires non conforme à nos standards. L’Union européenne interdit sur son sol les hormones de croissance depuis 1998 et, en théorie, l’importation de viande de bœuf et de volaille élevés avec ces produits. Mais, faute de traçabilité et de contrôle suffisants, Bruxelles ne peut pas garantir que la viande importée respecte ces obligations. De la même manière, les antibiotiques de croissance sont interdits dans l’Union européenne depuis 2006, mais aucune réciprocité ne s’applique. Face à ces réalités, les avantages économiques présumés de l’accord ne peuvent pas être invoqués. Selon la dernière analyse commandée par la Commission européenne,

Bien que cet accord ne nous soit pas profitable en l’état, nous ne pouvons pas non plus en faire une généralité et condamner ainsi tous les accords de libre échange, comme je l’ai entendu à l’instant. Les accords nous ont permis de croître et de faire rayonner hier et aujourd’hui nos produits, nos savoir faire dans le monde entier.

il est indéniable que l’ouverture d’un marché représentant 300 millions de consommateurs et 80 % du PIB de l’Amérique latine peut être une chance pour nos producteurs. C’est vrai pour nos spiritueux, pour nos produits laitiers ou encore pour notre industrie automobile. C’est pourquoi nous devons continuer à négocier pour inscrire dans ce contexte nos critères sanitaires et environnementaux, ainsi que les clauses miroirs indispensables. Si l’accord venait à être signé en l’état, malgré l’opposition résolue de la France, cela marquerait un tournant important pour notre pays en Europe. À l’inverse, le dossier a également valeur de test pour le futur de la politique de libre échange de l’Union européenne alors même que le Commission entame son nouveau mandat. Il sera regardé de très près par les autres pays avec lesquels l’Union négocie les accords commerciaux. Nous sommes ainsi face à une question purement politique, et non seulement économique et commerciale.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Mercosur étant en négociations depuis une vingtaine d’années, il m’est difficile de concevoir aujourd’hui la nécessité de se précipiter. Entre le mandat donné à l’Union européenne par les États membres et aujourd’hui, le cadre a beaucoup changé. L’inflation normative a multiplié les exigences pour nos agriculteurs en Europe, particulièrement en France. Nos normes environnementales et sanitaires européennes ont aussi beaucoup évolué. Nous ne pouvons pas non plus oublier le contexte national récent. Après les fortes mobilisations et manifestations agricoles du début d’année, l’imminence de la signature de l’accord remobilise les agriculteurs, exténués par le sentiment d’être encore une fois la variable d’ajustement. Le volet agricole inquiète particulièrement en France, car la ferme France n’est plus aussi compétitive. De deuxième exportateur mondial de produits agricoles au début des années 2000, la France a dégringolé et se situe avec une balance commerciale qui se dégrade fortement depuis. Ce débat sur le Mercosur nous invite inévitablement à nous questionner, sur les conséquences, entre autres, de surtranspositions européennes en France. Nous avons voulu aller vite, très vite, trop vite pour l’environnement et la santé.

Nos contraintes sont plus lourdes que celles de nos voisins. Il est urgent d’aligner les normes françaises sur les normes européennes, afin d’éviter toute distorsion de concurrence interne à l’Union européenne et de pouvoir enfin discuter de ce traité commercial de manière cohérente avec nos alliés européens. Jusqu’alors fierté nationale, notre agriculture semble aujourd’hui déconsidérée. Le Mercosur n’en est pas la cause, mais il pourrait briser un peu plus encore la compétitivité de notre agriculture française.

Or nos normes sanitaires et environnementales sont aux antipodes : antibiotiques, agriculture intensive, faible traçabilité, déforestation, utilisation de pesticides interdits, etc. Nous ne pouvons pas enclencher une telle marche arrière. La suppression de la majorité des droits de douane fait dès lors craindre une déstabilisation de certaines de nos filières agricoles européennes face à cette concurrence déloyale, car nous ne nous jouons pas avec les mêmes règles. La signature de cet accord en l’état aurait des conséquences sur nos filières de viande bovine, de sucre ou encore de volaille, et fragiliserait nos exploitations, qui n’ont réellement pas besoin de cela en ce moment. moment. Nous entendons que certains aspects de cet accord pourraient offrir des possibilités, y compris pour certaines filières agricoles. Le vin, les spiritueux, le fromage pourraient en tirer profit. C’est également le cas d’autres secteurs et services à forte valeur ajoutée, comme la chimie, les produits pharmaceutiques ou encore l’automobile. Un accord de libre échange facilitera l’import de métaux rares, indispensables aussi à nos économies pour l’électronique, le numérique et même les voitures électriques. Les crises de ces dernières années, climatique, sanitaire ou liée à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, de même que les tensions géopolitiques actuelles et la menace d’une nouvelle guerre commerciale avec la Chine et les États Unis nous incitent à diversifier nos partenariats. Aujourd’hui, trouver de nouveaux débouchés pour notre économie, limiter notre dépendance économique à quelques acteurs, trouver des solutions pour le secteur stratégique est, certes, nécessaire pour pouvoir résister aux menaces extérieures.

et nous ne voulons ni sacrifier notre agriculture et nos agriculteurs, qui sont un des joyaux de notre pays, ni transiger sur nos ambitions environnementales. Le commerce international peut se révéler une chance, pour peu que les règles du jeu soient équitables. Aujourd’hui, nous entendons l’inquiétude de nos agriculteurs. Nous ne sommes pas favorables à ce jour à un accord avec les pays du Mercosur, en tout Nous avons besoin de réassurances sur différents aspects. Nous devons ainsi nous donner les moyens de réaliser de manière régulière les contrôles sanitaires existants et renforcer la traçabilité et avoir réellement la possibilité d’activer la clause de sauvegarde en cas de besoin.

Ces points sont déterminants. Nous comptons sur la France et sur ses partenaires européens pour lever nos inquiétudes et trouver une solution équilibrée, sans nous diviser.

Nous souhaitons que se poursuivent les travaux entre l’Union européenne et le Mercosur et nous voulons être rassurés sur nos demandes, qui sont indispensables. Nous ne pouvons pas, en l’état, soutenir la position de la Commission européenne. Il y va de notre souveraineté alimentaire.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous félicitons de la tenue de ce débat consacré au traité de libre échange avec le Mercosur. Depuis vingt cinq ans, des négociations sont menées, dans l’opacité la plus totale, à l’abri des regards et des délibérations des peuples et des parlements nationaux, de part et d’autre de l’Atlantique. Pis, la Commission européenne voudrait désormais scinder le texte pour permettre l’exécution provisoire de son volet commercial, soustrayant ainsi sa mise en œuvre aux votes des assemblées des États membres.

Chers collègues de la droite sénatoriale, maintenant que certains d’entre vous sont devenus ministres, il serait temps de laisser l’Assemblée nationale se prononcer avons voté. Nous partageons les inquiétudes des syndicats agricoles, des ONG et des peuples mobilisés unanimement contre cet accord avec le Mercosur. Les exploitations sud américaines peuvent fournir des stocks d’importation sans équivalence possible pour l’agriculture française et européenne. Si l’on ajoute ces quotas à ceux qui sont prévus par les dix sept autres traités de libre échange en cours, on fera face à un véritable social et environnemental et à une mise en concurrence déloyale entre des systèmes de production très différents. Comment un éleveur de charolaises ou de limousines pourra t il rivaliser demain face aux éleveurs de bœufs sud américains, mais aussi canadiens, néo zélandais et de beaucoup d’autres pays ? Ce sera impossible L’aboutissement de ce traité empêcherait l’Europe de travailler à un nouveau pacte agricole, à une meilleure rémunération des paysans et à une alimentation de qualité accessible.

le secteur agro industriel prive déjà de terres près de quatre millions de petits paysans et multiplie les atteintes aux droits des populations autochtones. Et la question sociale n’est pas la seule qui se pose. La finalisation de cet accord entraînerait également des effets dramatiques sur le climat. Pour les pays du Mercosur, il promeut un système de monoculture intensif, nocif pour nos sols, la biodiversité, l’Amazonie et la stabilisation du climat. Il entraînera, des flux renforcés, une hausse de plus de 5 millions de tonnes des émissions de gaz à effet de serre, en favorisant le commerce de biens polluants, telles les voitures thermiques, interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Souhaitons nous réduire notre impact environnemental afin de garantir aux futures générations une planète habitable ou ne cherche t on finalement qu’à délocaliser notre pollution hors d’Europe ? Il en va de même pour l’exportation de produits chimiques, notamment des pesticides interdits en Europe. Chers collègues, comment justifier l’interdiction, légitime, de ces substances, qui contraint nos agriculteurs à modifier leurs pratiques pour protéger notre santé à toutes et tous, si elles sont autorisées dans les produits alimentaires importés ? Une mesure générale doit être prise d’urgence : l’interdiction des produits importés qui ne répondent pas à nos normes sociales et environnementales. Les prétendus gains de pouvoir d’achat ne peuvent pas être obtenus au détriment

somnifères qui permettent d’imposer la mise en œuvre à marche forcée de ce type d’accord. L’entrée en vigueur de nouvelles exigences est trop incertaine, notamment si l’on tient compte de la situation géopolitique.

Près de trois cents petits producteurs sont d’ores et déjà laissés sur le carreau. Quel modèle agricole européen voulons nous et, au delà, quel modèle de développement humain ? Souhaitons nous répondre aux besoins de la population ou permettre aux groupes agro industriels d’accroître leurs bénéfices en produisant là bas pour réimporter ici ? Si Emmanuel Macron a fait part de son opposition à l’aboutissement des négociations, pourquoi le mandat de négociation français n’a t il pas été révoqué ? N’est ce pas une opposition de façade ?

pour aboutir d’une opacité totale. Il protège non pas les peuples, mais les profits des multinationales européennes, qui cherchent de nouveaux débouchés, à l’heure où les États Unis développent un protectionnisme agressif contre nos industries. Pour notre part, nous refusons d’aggraver ce système de prédation fondé sur l’appropriation des fruits du travail et sur des discriminations systémiques envers les femmes, les autochtones et les travailleurs étrangers. À la violence de la libre circulation des capitaux et des marchandises, nous préférons un nouveau type de coopération avec les peuples du Mercosur, qui commencerait par la reconnaissance et la réparation de la dette coloniale que nombre de pays européens ont creusée dans ces pays. Tout rapprochement devrait être fondé sur les valeurs de solidarité, d’égalité et d’équité, et déboucher sur des investissements vertueux participant à l’indispensable bifurcation environnementale, afin de garantir une bonne vie pour toutes et tous, de chaque côté de l’Atlantique.

à une époque où l’on parlait peu du dérèglement climatique, des pollutions chimiques, de l’explosion des cancers, de la malbouffe ou encore de la souffrance animale. Il a été conçu à une époque où les gouvernements assumaient d’abandonner les classes populaires ici pour les exploiter là bas, de l’autre côté de la planète, et assumaient de faire de chaque hectare de terre, et bientôt de chaque parcelle d’intimité, une marchandise à vendre, à exploiter, sur le seul critère de sa rentabilité.

plus de 200 000 fermes ont aussi disparu dans notre pays. Cet accord, c’est la mondialisation du dérèglement climatique, de l’effondrement de la biodiversité et de l’extinction des espèces

D’ailleurs, lorsque Bolsonaro était au pouvoir, il n’a pas simplement incendié l’Amazonie au service de l’agrobusiness du soja et de la viande, il a aussi autorisé de nombreux pesticides extrêmement dangereux.

n’est pas un concept cynique et mercantiliste. Nous n’avons ni le fantasme d’une agriculture française qui nourrirait la planète ni celui d’une compétitivité acquise à coups de subventions publiques, au mépris des revenus des paysans, de l’environnement, de la santé, des territoires, des terroirs et de l’alimentation. La souveraineté alimentaire que nous défendons depuis les années 1990, c’est le droit pour un pays ou pour une communauté de pays de décider démocratiquement de l’organisation de son agriculture et de son alimentation, notamment pour éviter de dépendre excessivement de l’extérieur, y compris pour les intrants, les pesticides et autres semences. Pour nous, la souveraineté alimentaire revient à privilégier systématiquement les producteurs, les consommateurs et les citoyens au détriment – c’est très clair – de l’agro industrie, de l’agroalimentaire et de l’agrochimie. chers collègues, notre dernier enjeu de cohérence est celui du choix de notre modèle agricole. On ne peut pas refuser un jour les importations au nom d’une agriculture européenne plus vertueuse pour en sacrifier le lendemain les vertus. En arrivant au pouvoir, Bolsonaro et Trump ont directement attaqué les agences publiques chargées de la protection du climat, de la santé et de la biodiversité. Je regrette pour ma part très sérieusement les discours et les propositions

Merci

économique et commercial global (Ceta), ce projet d’accord soulève des inquiétudes quant aux répercussions à la fois économiques et sanitaires des nouveaux contingents qui seront autorisés à pénétrer le marché européen.

Dans le nouveau cadre d’échanges, l’Union européenne s’engage à abaisser ses barrières tarifaires sur la viande bovine, la volaille, le sucre et l’éthanol. Quelque 160 000 tonnes de viande bovine, principalement des morceaux à haute valeur ajoutée,

Alors que l’Union européenne défend et impose une agriculture vertueuse sur le plan environnemental et sanitaire nécessitant des investissements coûteux, Bruxelles laisserait entrer dans le même temps des produits agricoles sud américains, à rebours de ses propres prescriptions.

Ils n’ont pas peur de la compétitivité – je l’ai déjà dit à cette tribune –, à la condition que les mêmes règles s’imposent à tous. Dans la perspective d’autres accords potentiels avec le Mexique, le Chili, l’Inde, le Kenya, l’Indonésie ou encore la Thaïlande, la construction d’un régime solide de clauses miroirs est une nécessité absolue. Je rappellerai les propos de l’ancien président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, dans son discours du 13 septembre 2017 sur l’état de l’Union : « L’Europe est ouverte au commerce, oui. Mais réciprocité il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons. Sept ans plus tard, l’Europe s’est oubliée. Elle est divisée, sans stratégie commune, privilégiant des postures individuelles sous couvert d’une industrialisation en perte de vitesse, qui la pousse à abandonner ses agriculteurs et pose la question de notre souveraineté alimentaire qui s’érode.

la déforestation repousse souvent sur des terres montagneuses moins fertiles les populations et les petites structures agricoles au profit des plus puissantes. En Colombie par exemple, l’accaparement des terres au profit d’une dizaine de familles s’est développé après la signature du traité de libre échange entre l’Union européenne et la Colombie, qui s’applique depuis 2013. Résultat, les exportations se font au détriment du marché intérieur et de l’agroécologie paysanne. Enfin, l’accord de libre échange avec le Mercosur constitue un enjeu démocratique. Pour contourner la position de la France, qui pourrait faire valoir son droit de veto dans le cadre de l’approbation d’un accord mixte, la commission pourrait procéder à une scission du texte pour en extraire un accord commercial relevant exclusivement de la compétence de l’Union européenne. Ce projet porterait atteinte aux parlements nationaux. Il ne respecterait pas le mandat de négociation initial donné par le Conseil européen à la Commission. Il serait très inquiétant pour l’avenir de l’Europe que la confiance soit ainsi bafouée d’un simple revers de main. Rappelons qu’à la signature de l’accord d’association entre la Commission européenne et le Mercosur, le communiqué du 28 juin 2019 de la commission était clair Le nouveau cadre commercial, composante d’un accord d’association plus large entre les deux régions, consolidera un partenariat politique et économique stratégique et offrira d’importantes possibilités de croissance durable à chacune des parties, tout en respectant l’environnement et en préservant les intérêts des consommateurs et des secteurs économiques sensibles de l’Union européenne.

La France doit rester ferme. Elle ne cédera pas aux arrangements entre faux amis. Nous continuerons le combat pour que cet accord ne voie pas le jour

mes chers collègues, tout cela n’est finalement que le symptôme de la profonde obsolescence d’un système de libre échange qui a ravagé conjointement l’environnement et nos économies. Le Mercosur n’est que le dernier avatar de cette conception uniquement comptable de l’homme et des économies il n’y aurait que flux, échanges et avantages comparatifs à faire se rencontrer, au mépris complet des espaces, de la biodiversité et de nos agriculteurs, le tout pour surseoir quelque temps à l’agonie de l’industrie allemande.

Il y aurait ainsi d’un côté les mauvais traités de libre échange, qui détruisent nos entreprises et nos agricultures, qui ravagent les paysages et le climat, et font vendre à des chômeurs des biens produits par des esclaves ; et il y aurait de l’autre côté

la compétence exclusive de l’Union européenne sur les négociations commerciales. La voix de la France, la voix de son Parlement, la voix des Français, tout cela est sans effet sur les pouvoirs que s’est arrogés la Commission. Le Rassemblement national se félicite d’avoir été constant, non pas dans l’opposition à l’Europe que nous défendons comme ensemble culturel et civilisationnel, mais à cette construction européenne qui s’est

Monsieur le sénateur Didier Marie, vous avez rappelé que céder, c’était renoncer à la capacité de régulation. Je crois personnellement à la capacité de régulation de l’Union européenne.

! Monsieur le sénateur Patriat, vous avez eu raison de dire à quel point notre agriculture était notre fierté. Vous avez aussi fait la démonstration éclairante de l’effet de l’importation de certaines productions, par exemple en viande bovine,

Monsieur le sénateur Menonville, vous avez à juste titre rappelé à quel point les garanties environnementales avaient été rehaussées dans l’Union européenne.

conclus à n’importe quel prix et en tout cas pas au prix du sacrifice de nos agriculteurs et de notre agriculture. La parole

à redoubler de protectionnisme et à soutenir leurs filières agricoles et leurs secteurs industriels face aux intérêts européens. Nous ne pouvons pas être les derniers naïfs

Ce vote illustre notre volonté commune de préserver les principes fondamentaux de solidarité républicaine et d’égalité territoriale. En maintenant un tarif figé équitable pour les trajets entre la France hexagonale et les territoires ultramarins, nous reconnaissons les réalités spécifiques de ces territoires, où le transport aérien est non pas un luxe, mais une nécessité vitale. Cette mesure corrige une iniquité tarifaire qui pesait particulièrement sur les populations déjà confrontées à des défis économiques majeurs. Les déplacements professionnels, médicaux ou familiaux sont indispensables et augmenter leur coût reviendrait à accroître encore les inégalités. Il était donc de notre devoir d’agir pour garantir une mobilité accessible et équitable à tous nos compatriotes. Cette décision dépasse la seule question économique. Elle représente un geste fort envers des populations qui se sentent souvent éloignées des décisions prises ici, dans l’Hexagone. En adoptant ce sous amendement, nous affirmons notre volonté de renforcer le lien indéfectible qui unit la République à ces territoires ultramarins. Encore une fois, je vous remercie pour cet engagement collectif en faveur de la justice et de l’équité.

que nous augmentions progressivement et chaque année les taux d’incorporation de biocarburants dans les carburants d’origine fossile. En effet, les biocarburants constituent une solution de remplacement crédible, notamment pour les poids lourds,

du Gouvernement ? La modification des paramètres de la Tiruert, en dehors des tarifs, doit être prévue au minimum une année en avance afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux objectifs fixés. Une hausse trop importante des objectifs en la matière pourrait déstabiliser le marché. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

seront éligibles à la déduction fiscale. Ces carburants doivent être embarqués en France pour des vols depuis la France vers des destinations extracommunautaires. Un décret fixera les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul du crédit d’impôt, ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises éligibles. la somme des crédits d’impôt ne pourra excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice. Nous devons montrer que nous ne sommes pas uniquement dans une logique

durables entre 2025 et 2050, échéance au delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs. Pour atteindre cet objectif ambitieux, c’est toute une filière

est à M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxe sur le kérosène pour les vols commerciaux effectués en jets privés et pour les vols intérieurs.

Pour une installation moyenne de 5 000 euros, le surcoût s’élèverait à 725 euros, soit une somme considérable, en particulier pour les foyers modestes.

en contradiction avec l’objectif affiché de ne pas alourdir l’imposition des classes modestes et moyennes. Elle s’éloigne significativement du taux de 10 % initialement proposé par le Gouvernement et risque de freiner la nécessaire modernisation du parc de chauffage Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article

Cet amendement vise à rétablir le bénéfice de la TVA à taux réduit pour le remplacement d’une chaudière susceptible d’utiliser des énergies fossiles. Si nous ne remettons pas en cause la nécessité de sortir des énergies fossiles,

en plus de la chaleur, l’électricité utilisée pour faire fonctionner ces réseaux.

le développement de l’ensemble des modalités de production de chaleur et de froid géothermiques en appliquant le taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des composantes de la fourniture d’électricité,

actuellement le taux de 20 %. Si la géothermie est aujourd’hui bien identifiée comme un levier incontournable de la transition énergétique, elle est encore, hélas ! largement sous utilisée. À ce jour, les solutions géothermiques ne représentent que 1 % de la consommation finale de chaleur et 5 de l’énergie entrante des réseaux de chaleur en France métropolitaine, tandis que la stratégie française de transition énergétique prévoit de multiplier par trois la production de chaleur géothermique d’ici à 2035. Le coût de l’électricité nécessaire au fonctionnement des installations géothermiques représente une part non négligeable de leurs coûts d’exploitation. Des taux réduits de TVA permettraient de renforcer la compétitivité de la géothermie et d’accompagner l’essor de la filière en France, absolument indispensable pour poursuivre la décarbonation des usages grâce à une énergie locale,

en particulier en matière de décarbonation de la production de chaleur et de réduction de l’importation d’énergies fossiles. La valorisation énergétique des déchets représente par exemple la première source de production de chaleur vertueuse dans nombre de nos territoires. Nous souhaitons tous continuer d’étendre